d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie en début d'après-midi, sont consultables sur le site du Sénat.

Le décret du 14 mai 2020 prévoit l'attribution d'une prime aux professionnels des établissements publics de santé, qui ont mobilisé toutes leurs forces pour vaincre l'épidémie de coronavirus. Il a suscité de vives réactions de la part des personnels soignants, tant il est injuste et inéquitable dans son application, le montant de cette prime variant de 500 à 1 500 euros selon l'établissement ou la situation géographique. cette distinction est très mal vécue par les personnels concernés, qui y voient un manque de reconnaissance de la Nation pour leur action, leur engagement pourtant sans faille, sans compter que certaines professions sont exclues de ce dispositif de prime. C'est le cas, par exemple, des aides à domicile, qui ont, malgré la quasi-absence d'équipements de protection individuelle au départ, continué à assumer pleinement leur rôle, en première ligne auprès des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap. Elles ont notamment aidé nos concitoyens les plus vulnérables à supporter l'isolement pendant le confinement. Ce sont ainsi 300 000 professionnels de l'aide à domicile qui sont exclus du bénéfice de Toutes les professions exposées au virus doivent être récompensées par la Nation. Or le Gouvernement a pris la décision de ne verser des primes qu'aux personnels d'État de la santé et du médico-social, laissant notamment aux collectivités locales le soin d'assumer les dépenses pour certains autres professionnels. Dans le contexte que nous connaissons, cela n'est pas acceptable ! Ma question est simple : que comptez-vous faire pour tenir vos promesses et garantir une équité de traitement entre tous les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social ?

sans attendre les changements profonds qui feront suite au « Ségur de la santé », cette concertation historique qui aboutira, nous l'espérons tous, aux accords de la santé, nous avons en effet décidé de verser une prime exceptionnelle aux professionnels qui ont permis au système de santé de prendre en charge un afflux majeur de patients contaminés par le Covid-19.

Tous les soignants mobilisés pendant la crise sanitaire bénéficient d'une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, quel que soit leur statut, public ou privé, ou leur activité. Dans les quarante départements les plus touchés par l'épidémie, cette prime est majorée et s'élève à 1 500 euros. Dans ces départements, ce sont un peu plus d'un demi-million d'hospitaliers qui percevront cette prime. Dans les autres départements, la prime s'élèvera à 500 euros au sein des services hospitaliers les plus mobilisés dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Le directeur de l'établissement peut d'ores et déjà relever le montant de la prime à son maximum pour les services ou les agents les plus impliqués dans la prise en charge de patients contaminés.

l'assurance maladie prend en charge le versement de la prime pour tous les établissements et services tarifés par l'assurance maladie, y compris lorsque celle-ci n'est pas tarificateur unique. Ce mécanisme conduit des services de soins infirmiers à domicile

les casseurs et la délinquance ; les policiers et les gendarmes assurent jour et nuit le maintien de l'ordre, souvent au péril de leur vie. C'est dire à quel point est malvenue la campagne contre les violences policières menée par des identitaires racialistes, dont l'idéologie et les objectifs sont à l'opposé de l'antiracisme qu'ils font mine de professer. Cette campagne vise à imposer une grille de lecture américaine sur la situation française, qui n'a pourtant rien à voir. Une grande majorité de nos concitoyens en sont choqués et refusent les antagonismes suscités par ceux que le Président de la République a appelés les « séparatistes ». La vérité est que l'immense majorité des violences que constatent les Français portent atteinte à l'ordre républicain les guets-apens tendus aux forces de sécurité, les trafics de drogue, l'incroyable guerre des gangs qui vient d'avoir lieu à Dijon. Dans ces conditions, les discours scandaleux de certains agitateurs bien connus, pleins d'arrière-pensées, qui portent atteinte à la réputation des policiers et des gendarmes sont plus qu'inconvenants. La police française n'est pas raciste, et ses membres acceptent pleinement que les fautes de certains soient sanctionnées, car c'est la condition de leur exemplarité. Les forces de l'ordre doivent savoir qu'elles bénéficient de l'entier soutien des institutions de la République, de leurs autorités de tutelle et de la très grande majorité du peuple français. Monsieur le ministre, les syndicats de policiers demandent que vous réarmiez la police juridiquement, moralement et matériellement. Comment comptez-vous faire ?

chaque jour, chaque nuit, à chaque instant, la police et la gendarmerie interviennent sur nos territoires, urbains comme ruraux, dans des moments de tension, dans le quotidien, pour protéger les Français. Trop souvent, en effet, ils doivent faire face à des provocations, à des insinuations, à des menaces, à des injures et à des mises en cause incessantes.

droit. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, la société française va mal,

et de vivre ensemble, de construire quelque chose ensemble ? Faire nation, ce n'est pas simplement considérer le passé pour ce qu'il est, c'est construire à partir de ce passé, c'est imaginer où nous voulons aboutir en tant que peuple. Or, de ce point de vue, nous avons manifestement une difficulté à nous projeter. Certains remettent explicitement en cause les fondements du pacte républicain.

le respecter ; c'est parce qu'il est l'émanation de notre Nation et parce qu'il est là pour faire respecter un certain nombre de règles essentielles à l'intérêt commun.

Il faut soutenir ceux qui mènent le combat de la République. Le ministre de l'intérieur a ainsi mille fois raison de soutenir les forces de l'ordre. Elles sont au coeur de ce combat pour la République, mais elles ne sont pas seules

L'État est aussi le garant de l'unité de la Nation, et lorsque la société est de plus en plus violente et de plus en plus fracturée, il faut s'appuyer pleinement sur ceux qui défendent la République.

terribles événements qui ont secoué des quartiers de Dijon et de Chenôve ces derniers jours. Je voudrais d'abord souligner la présence de M. le secrétaire d'État Laurent Nunez hier à Dijon. Sa venue était essentielle après quatre jours de violences urbaines

elle était attendue aussi par les forces de l'ordre et les services préfectoraux, qui ont, avec les moyens disponibles et beaucoup de sang-froid, contenu une situation sans précédent. Vous avez annoncé des effectifs supplémentaires pour assurer le maintien de l'ordre et réaffirmé la détermination de l'État à poursuivre les auteurs des faits et à les sanctionner. Cela devait être fait.

Pourquoi a-t-il fallu attendre trois jours avant que des renforts ne soient effectivement affectés ? Enfin, plus globalement, monsieur le ministre, face au développement de telles violences et au besoin de sécurité de nos populations, comment pensez-vous faire évoluer l'organisation et les moyens des forces de l'ordre ? La

de ce groupe d'individus dans la ville de Dijon n'avait pas été anticipée en matière de renseignement. Pourtant, les forces de sécurité intérieure, qui n'étaient pas numériquement en mesure de faire face et n'étaient pas préparées, ont répondu présent.

comme vous, je refuse que la crise puisse alimenter une fracture entre générations. J'ai été frappé par certains discours qu'on a pu entendre pendant cette crise, présentant les jeunes comme un risque et les personnes âgées comme un poids.

plan de relance pour la jeunesse. Il ne s'agit pas uniquement de protéger la jeunesse des risques économiques, mais bien, comme vous l'avez dit, de la placer au coeur de la relance. En effet, les entreprises et les secteurs d'activité d'avenir sur lesquels nous allons parier auront besoin de la créativité et de la mobilisation des jeunes pour relever le pays.

Ils sont 800 000 à s'apprêter à entrer dans la vie active, mais ils craignent d'être une génération sacrifiée, la variable d'ajustement d'un marché de l'emploi totalement déstructuré. Les difficultés économiques qui touchent nombre de nos TPE et PME, qui sont les premiers employeurs, par contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, de notre pays, fragilisent ces voies d'insertion professionnelle.

Il faut donc assortir ces aides d'une promesse de contrats plus sécurisants. Il faut également que les entreprises puissent bénéficier des mêmes aides quand elles concluent des contrats de professionnalisation Enfin, celles qui parviendront à embaucher nos jeunes de moins de 30 ans des contrats plus classiques doivent pouvoir bénéficier de l'exonération des charges. Il faut aussi lever les freins à l'embauche par des mesures complémentaires de celles concernant l'emploi. Je pense notamment à l'examen du permis de conduire. J'ai écrit vendredi au ministre de l'intérieur pour l'alerter sur la situation catastrophique qui se profile dans plusieurs départements. En Gironde, le confinement a créé un stock de plus de 6 000 examens en attente,

Les jeunes ne peuvent pas passer le permis en temps et en heure, et ils le paient ! Madame la ministre, si nous ne pouvons pas nous serrer la main, nous devons du moins nous serrer les coudes pour nos enfants et construire avec l'ensemble des partenaires de l'emploi un plan ambitieux pour l'insertion professionnelle des jeunes. Le temps presse

un grave risque, compte tenu de la crise économique et sociale qui suit la crise sanitaire. Un pays qui n'investit plus pour sa jeunesse n'investit plus dans son avenir.

Le Président de la République a déclaré dimanche dernier, lors de son allocution télévisée, qu'il fallait « bâtir un modèle économique durable, plus fort », travailler et produire davantage ». Le propos mériterait d'être éclairci, à l'heure où des centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi, sachant qu'autant vont subir le même sort dans les semaines à venir. « Travailler plus pour gagner plus » n'est pas une idée neuve pour un nouveau monde, puisque le concept fut créé par Nicolas Sarkozy. « Travailler plus » est l'objectif

Les premières victimes de votre politique sont les salariés peu diplômés et les jeunes, déjà durement touchés par les conséquences du confinement. Pourquoi vous obstinez-vous dans ces choix archaïques qui n'ont pas donné de résultats probants, sauf pour les actionnaires ? Quand allez-vous faire le choix d'une économie orientée vers l'emploi, au service d'une autre production, qui protège et qui donne du travail au plus grand nombre ? Allez-vous enfin partager le travail pour permettre l'épanouissement de chacun et cesser de contraindre toujours plus ceux qui ont un emploi tout en précarisant les autres ?

Cette mobilisation pour que tout le monde puisse travailler, et vite, sera essentielle pour maintenir l'activité : l'activité, c'est l'emploi ! Telle est la dynamique que nous voulons favoriser très rapidement : il ne faut pas attendre, car l'emploi n'attendra pas

permettrait le travail de toutes et de tous. La France, dont la productivité est l'une des plus fortes au monde, en a les moyens ! Quelle société voulons-nous : celle de la précarité et du chômage de masse, ou celle qui permet à tout le monde de travailler ? La

Refusant de faire nation, des minorités hystérisées veulent récrire l'histoire de France. On macule la statue du général de Gaulle. On appelle à déboulonner Louis XIV, Napoléon, Jules Ferry. On crache sur les figures qui ont bâti notre histoire. Des tentations obscurantistes guettent notre société. Certes, dimanche dernier, le chef de l'État a condamné une « réécriture haineuse ou fausse ». « On ne déboulonnera pas de statues », a-t-il martelé. Ces propos effacent-ils pour autant ceux du candidat qu'il fut, déclarait que la colonisation était un crime contre l'humanité, une vraie barbarie pour laquelle il devait présenter ses excuses ? Sous le buste de Jean-Baptiste Colbert, grand commis d'État qui fit de notre pays une puissance navale, sous les auspices de Jules Ferry, qui présida notre assemblée et fonda notre école républicaine, Premier ministre, que les travaux historiques et scientifiques, qui replacent toujours l'action des femmes et des hommes dans leur époque, seront protégés ? Êtes-vous prêt à ne jamais laisser récrire l'histoire, à ne jamais laisser faire le tri entre faire le tri entre zones d'ombre et passages étincelants au gré des émotions du moment ? Pouvez-vous nous assurer que l'on continuera à écrire et à enseigner l'histoire de France, non sous la dictature d'une pensée militante et largement communautariste, mais avec l'esprit civique et critique et la recherche de l'universalisme qui caractérisent l'héritage des Lumières

qui suivirent. Nous sommes au Sénat, haut lieu de la République, mais nous travaillons sous les auspices de Saint Louis, parce que c'est l'histoire de la France !

Monsieur le Premier ministre, je vous ai demandé de protéger les travaux des historiens et la possibilité pour eux d'écrire l'histoire avec l'esprit critique qui nous caractérise. Marc Bloch rappelait que, entre tous les péchés, au regard d'une science du temps, le plus impardonnable était l'anachronisme. Or c'est bien l'anachronisme qui anime aujourd'hui des minorités prêtes

La crise sanitaire a entraîné une récession économique et sociale qui nous oblige à repenser nos modèles de consommation et de production. Alors que le manque de visibilité des plans de relance inquiète les entreprises et les salariés, entreprises et les salariés, de nombreuses voix s'élèvent pour demander que la sortie de crise de 2020 ne ressemble pas à celle de 2008, quand les programmes de soutien à l'économie avaient entraîné une hausse significative des émissions de CO2. Certes, il faut rapidement soutenir la reprise d'activité et relancer l'emploi, mais ignorer l'impérative nécessité de construire, dès aujourd'hui, le projet d'une économie verte serait nous devons soutenir dans l'urgence les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile, mais il faut mobiliser, dès maintenant, des aides financières significatives et vite engager une réflexion sur la formation des salariés à de nouveaux métiers pour réussir le verdissement de la production. Or Airbus envisage de couper dans son budget de recherche et développement, alors même que, dans la course à l'hydrogène, l'Allemagne n'a pas attendu pour investir massivement dans l'hydrogène vert. De même, nous devons construire une politique volontariste de rénovation thermique des bâtiments et des logements : Mme la ministre de la transition écologique l'appelle de ses voeux et le secteur du bâtiment est prêt à la mettre en oeuvre.

conclusion, la transition écologique et énergétique sera très clairement au coeur du plan de relance que nous allons mettre en oeuvre. Nous ferons des annonces fortes. Le Président de la République a tracé le chemin. Que ce soit en matière de rénovation thermique, de mobilités vertes ou d'investissements au service de l'industrie décarbonée, nous serons au rendez-vous

madame la ministre, mesurez-vous la gravité de la situation ? Des règlements de comptes en plein centre-ville, des bandes armées qui déferlent pour s'affronter avec une violence inédite et qui narguent la police et la justice : cela ne se déroule pas dans le chaos de pays lointains, mais bel et bien dans un quartier d'une paisible ville de province. L'État n'apparaît assurément plus assez fort pour y faire régner l'ordre public. La loi de la République est supplantée par la loi du plus fort et du plus violent. C'est la négation même de notre civilisation ; le tribalisme a remplacé la justice. L'impunité est devenue la règle ; les témoignages de policiers désespérés devant l'absence de peines ou le prononcé de peines symboliques se multiplient. Mais il y a pis encore que l'absence de peine ou la peine symbolique : vos récentes décisions, madame la ministre, constituent un véritable blanc-seing pour les voyous et autres délinquants.

Il y a deux façons de lutter contre la surpopulation des prisons : en construire de nouvelles- promesse du début du quinquennat passée aux oubliettes -ou vider celles qui existent, quitte à se laisser aller à l'injustice et à faire disparaître le sens même de la peine. Malheureusement, vous avez choisi cette seconde solution, qui s'accorde avec votre conception de la justice, hélas impuissante pour éviter l'embrasement du quartier des Grésilles. Vous préférez dicter aux juges le choix de la peine en fonction des capacités pénitentiaires. Quelle justice voulez-vous, madame la ministre ? Pensez-vous que le moment est bien choisi pour mettre en oeuvre la « régulation carcérale » que vous appelez de vos voeux, qui n'est ni plus ni moins que l'institutionnalisation d'une totale impunité ? Est-ce le moment de donner le signal que l'État baisse les bras ? Jusqu'à quel niveau de violence faudra-t-il aller avant que vous reconnaissiez faire fausse route ? Je vous invite, en conclusion, à méditer ces mots de Charles Péguy : « L'ordre, et l'ordre seul, fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude.

les mesures que nous avons adoptées pendant la crise sanitaire avaient une visée exclusivement sanitaire : il s'agissait d'éviter la diffusion du virus dans les milieux fermés que sont les prisons.

malgré les aides qui ont été annoncées. Il faut pourtant savoir qu'à cette période de l'année beaucoup de nos jeunes jouent leur avenir professionnel. Vous affirmez vouloir relancer l'industrie dans notre pays et y faire revenir des activités

Les métiers manuels n'attirent plus, alors que les artisans sont en demande. Ce type de formation ne doit plus être considéré comme une voie de garage lors de l'orientation scolaire. L'éducation nationale a un rôle immense à jouer pour que le collège oriente davantage vers les métiers manuels. Nos artisans ont façonné notre patrimoine, qu'il soit bâti, culinaire ou créatif. Pourtant, leurs métiers perdent peu à peu de leur attractivité, malgré les efforts des CFA et autres structures de formation. Nous devons revaloriser les CAP : combien de PME ont été créées par des hommes ou des femmes ne possédant que ce diplôme ? N'oublions pas que l'artisanat est la plus grande entreprise de France ! Cette crise a mis en difficulté toute notre économie. Les centres de formation s'inquiètent pour l'avenir : les entreprises seront-elles au rendez-vous ? Vous avez pris des mesures importantes importantes pour inciter les chefs d'entreprise à embaucher des apprentis ; je vous en remercie. Le Gouvernement va-t-il aider l'artisanat à retrouver la place qu'il mérite et développer les valeurs de l'apprentissage afin d'attirer les élèves vers des études manuelles ?

quoi qu'il vous en coûte, l'autorité de l'État est malmenée, malgré la brillante tirade de M. le Premier ministre en réponse à l'intervention édifiante de Roger Karoutchi. L'autorité républicaine est malmenée par la violence, par le mépris des forces de l'ordre, des forces de l'ordre, mais aussi par des comportements qui substituent la tambouille électorale au respect des principes démocratiques. Ce n'est pas la règle qui doit vous tenir ; c'est à vous de tenir la règle. Il n'y a de démocratie que si les élections se tiennent à des dates fixes et régulières. Alors que les élections régionales sont prévues au mois de mars 2021, les raisons annoncées d'un report de plus d'un an laissent perplexe, inaugurant la fixation de la date d'élections pour convenance personnelle, au mieux, pour convenance de La République En Marche, au pire. Selon la presse, le Président de la République, descendant du grenier à la cave, se serait livré à des tractations de marchands de tapis avec les présidents de région : « Je Je vous aide financièrement si vous m'aidez à reporter les régionales après la présidentielle, car j'ai des opposants politiques parmi vous. Je ne vais pas donner de l'argent à mes adversaires, On apprend que le Président de la République a des adversaires, et n'est donc pas le président de tous les Français, considérant que l'argent public des régions est le sien et que, du fait du prince, il peut le distribuer à qui bon lui semble. Comme le disait Xavier Bertrand, « derrière les élections, il y a le peuple, et le peuple, on le respecte ». Monsieur le ministre, allez-vous renoncer à cette manoeuvre grossière ? Allez-vous travailler avec toutes les régions élues démocratiquement et dont une compétence légitime est le développement économique ? La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

de discuter avec les présidents de région de la meilleure façon de les accompagner dans la mise en oeuvre concrète de leur action pour défendre l'économie de nos territoires et relancer l'emploi partout où c'est nécessaire,

Nombre de filières agricoles, partout dans notre pays, sont particulièrement touchées par la crise sanitaire et économique du Covid-19. Il conviendra d'ailleurs de tirer les leçons de cette crise pour retrouver ce que la FNSEA et bien d'autres appellent une souveraineté alimentaire solidaire, qui devra associer- c'est un préalable indispensable -tous les acteurs publics et privés et s'appuyer sur une logique d'alimentation durable et locale. Je sais que le Président de la République, le Gouvernement et vous-même, monsieur le ministre, en faites une priorité dans le cadre de la relance, placée sous le signe de la transition écologique.

au travers de mécanismes financiers et de dispositifs visant à passer au mieux cette épreuve. J'en veux pour preuve les décisions prises et les moyens mis en place en faveur de la pêche et de l'aquaculture, de la viticulture ou de l'horticulture. Monsieur le ministre, vous connaissez bien le département du Nord pour vous y être rendu à plusieurs reprises. Terre de labeur, c'est aussi un grenier d'abondance pour le pays tout entier.

surtout les femmes et les hommes de la deuxième ligne, les agricultrices et les agriculteurs qui ont travaillé sans relâche pour produire et alimenter nos concitoyens, les entreprises de l'agroalimentaire, les coopératives agricoles, les transformateurs

souffrent. Le Ségur de la santé doit permettre de répondre à ces difficultés. Le Président de la République a promis un système plus souple, plus simple, plus proche, revalorisant le collectif, le sens de l'équipe et l'initiative des professionnels.

les syndicats d'infirmiers n'étaient même pas conviés ... Le doute gagne de très nombreuses organisations syndicales, qui déplorent des sujets escamotés et craignent que les arbitrages ne soient déjà réalisés. Elles redoutent un simulacre de concertation destiné à calmer leur colère.

Si l'on ne rompt pas avec le fléau bureaucratique, la centralisation de la décision, le cloisonnement des structures, l'augmentation des salaires soulagera momentanément la douleur sans soigner le mal profond.

en termes d'autonomie, et que les inégalités scolaires sont fortement liées aux origines sociales. La crise sanitaire n'a rien arrangé : nous avons perdu beaucoup trop d'élèves. Certes, monsieur le ministre, la communication sur les vacances apprenantes va bon train, laissant croire que tout est sous contrôle, mais quelle sera l'ampleur de ce dispositif ? Touchera-t-il tous les élèves qu'il faudrait, que, dans le même temps, la mesure exceptionnelle du 22 mars dernier, consistant à accorder un crédit d'impôt de 50 % pour les cours privés à distance, permettait déjà aux familles aisées d'assurer un accompagnement de leurs enfants pendant le confinement ? L'école est gratuite et obligatoire, et elle doit le rester. Elle doit être la même pour tous et permettre à tout enfant de France de devenir ce qu'il peut

porte sur la rentrée scolaire de septembre, cruciale comme jamais. Quelle est votre stratégie face à l'urgence absolue ? Quelles dispositions spécifiques seront prises concrètement afin de remédier au creusement des inégalités scolaires et numériques intervenu durant la crise et de permettre à tous les jeunes en âge scolaire de reprendre le chemin de l'école sans souffrir de retards irrécupérables ? La parole

que nos élèves sont sur une voie de progrès, en particulier dans les territoires les plus en difficulté, où 300 000 enfants bénéficient du dispositif de dédoublement des classes de CP et de CE1. Ces mêmes 300 000 enfants ont pu retourner

faudra peut-être mettre l'accent sur l'autonomie, la confiance en soi et le développement cognitif des enfants, de façon qu'ils s'épanouissent le mieux possible. Nous

du projet de loi organique portant report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles (projet n°

La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires économiques a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique portant report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles

de la démocratie. Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, le jour même où le Gouvernement décidait de convoquer les électeurs pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain, il adoptait en conseil des ministres deux projets de loi : le premier prévoyait la prolongation du mandat des conseillers municipaux dans les communes où le renouvellement n'avait pas été complet le 15 mars dernier

que de ne pas délibérer de textes virtuels, hypothétiques, de ne pas légiférer à blanc quand il existe une autre manière

et je vais m'en tenir là. Je n'aurais pas abordé cette question si vous n'aviez pas vous-même, monsieur le ministre, souhaité faire une mise au point à l'occasion de votre propos introductif.

être élus à la date prévue. Nous avons accepté que leur élection soit reportée au mois de mai 2021. Par conséquent, pour reprendre une expression dont je ne suis pas l'auteur, mais dont les commentaires autorisés du Conseil constitutionnel ont validé l'utilisation, le corps électoral des six sénateurs représentant les Français établis hors de France renouvelables

qui, par lui-même, soulève des critiques d'un point de vue constitutionnel s'il n'est pas circonscrit au traitement du cas de force majeure auquel nous sommes confrontés.

Nous nous trouverions dans une assez grande confusion, qui porterait préjudice à la représentation des Français établis hors de France.

de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France est sans incidence aucune sur le périmètre du renouvellement partiel du Sénat et les conséquences que la Constitution y attache. Il est important

qui soit lui-même l'émanation de ces collectivités ; que, par suite, c'est à juste titre que le législateur organique a estimé que le report en mars 2008 des élections locales imposait de reporter également l'élection de la série A des sénateurs afin d'éviter que cette dernière ne soit désignée par un collège en majeure partie composée d'élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal

Enfin, le report du renouvellement du collège électoral fonde le report de l'élection sénatoriale concernée. Ces éléments nous incitent à suivre le Gouvernement et la commission des lois. Toutefois, je m'interroge sur le cas de la Guyane, mais aussi d'autres départements. En effet, même s'il faut bien souligner que la disposition en cause n'a pas encore été promulguée,

». Si le nombre de scrutins reportés était élevé, on se dirigerait vers la création de fait d'une troisième série. Se poserait aussi fatalement la question des conseillers départementaux élus en 2015, qui n'auraient jamais été appelés aux urnes sénatoriales.

postulat que le second tour des élections municipales ne pourrait pas se tenir au mois de juin 2020 en raison de la crise sanitaire, il est prévu de reporter l'élection des 178 sénateurs de la série 2.

Je me réjouis que le Gouvernement ait procédé à la réécriture de son texte par le biais de plusieurs amendements. Un avis du Conseil d'État aurait effectivement pu nous apporter un éclairage intéressant sur des points juridiques délicats. Il est dommage qu'il n'ait pas été saisi. saisi. Comme les élections consulaires n'auront pas lieu à l'échéance prévue, trois solutions pouvaient être envisagées pour l'organisation de l'élection des six sénateurs représentant les Français de l'étranger

La deuxième solution, très simple, est de prolonger d'un an le mandat de ces six sénateurs représentant les Français de l'étranger, afin de procéder au renouvellement de leur mandat à la date la plus proche possible de l'échéance normale, à savoir septembre 2020. La troisième solution, qui constitue une variante de la précédente, consisterait à reporter l'élection des six sénateurs représentant les Français de l'étranger jusqu'au renouvellement partiel suivant du Sénat, soit en septembre 2023. Le Gouvernement a estimé que les conseillers consulaires ne pourraient pas élire les six sénateurs représentant les Français établis hors de France renouvelables en septembre 2020. Il a donc proposé de prolonger d'un an les mandats de ces six sénateurs et de réduire à due concurrence ceux de leurs successeurs. Je me félicite que la commission ait retenu cette solution, tout en procédant tout en procédant à un aménagement ; elle a précisé la nouvelle échéance du mandat des six sénateurs renouvelables en septembre 2020 en la fixant à septembre 2021- ce qui paraît logique -, alors que le Gouvernement prévoyait de renvoyer cette question à un décret.

L'élection en 2021 de six sénateurs représentant les Français de l'étranger constituerait ainsi un ajustement non seulement provisoire et mesuré, mais également rigoureusement proportionné aux circonstances exceptionnelles qui le motivent. le motivent. Ses conséquences juridiques seraient les mêmes que celles d'élections partielles organisées entre deux renouvellements partiels du Sénat pour pourvoir un ou plusieurs sièges vacants.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après avoir examiné la semaine passée le projet de loi ordinaire relatif au report des élections consulaires, nous sommes aujourd'hui réunis pour étudier un projet de loi organique traitant du report de l'élection de sénateurs représentant les Français établis hors de France.

C'est dommage, car le travail du législateur aurait été plus efficace, et nos débats moins tronqués. Au fond, il n'est principalement question, dans ces textes, que du report des élections consulaires et de ses conséquences. ses conséquences. Initialement, ces deux projets de loi avaient une portée bien plus large et plus virtuelle. Le Gouvernement souhaitait en effet qu'un certain nombre de modifications législatives soient adoptées « au cas où » le second tour des élections municipales n'aurait pas lieu le 28 juin prochain.

Reporter d'un an l'élection de l'intégralité des sénateurs de la série 2 ou seulement celle de six sénateurs représentant les Français établis hors de France, ce n'est pas la même chose. Il était nécessaire de bien mesurer les conséquences juridiques d'une telle modification ou, plus précisément, d'en analyser la constitutionnalité. Devons-nous reporter l'élection de ces six sénateurs, qui devait avoir lieu en septembre prochain ? Telle est donc la question que nous devons trancher aujourd'hui.

Ce dernier estime en effet depuis 2005 qu'il n'est pas possible, pour des élus dont le mandat a été prorogé- c'est, en l'espèce, le cas des conseillers consulaires -, de désigner durant cette prorogation de nouveaux sénateurs. Nous soutenons donc les modifications apportées au projet de loi organique par notre commission des lois, qui a choisi de reporter cette élection après les prochaines élections consulaires, en septembre 2021. solution pragmatique et efficace, qui permettra l'élection des sénateurs concernés dès que leur collège électoral aura été renouvelé. Leur mandat sera limité à cinq ans, afin de ne pas bouleverser durablement le calendrier électoral.

le reste du calendrier sénatorial demeurant inchangé. Le groupe Union Centriste soutiendra ce projet de loi organique dans la rédaction issue des travaux de notre commission des lois.

À nos yeux, le plus simple et le plus logique serait que l'élection des six sénateurs représentant les Français établis hors de France ait lieu au mois de septembre 2020, en même temps que celle de tous les autres sénateurs de la série

terme normal ». Or si l'on permettait aux conseillers consulaires en place de voter une nouvelle fois

serait donc pas contradictoire avec la lettre ni avec l'esprit de la décision du Conseil constitutionnel du 15 décembre 2005.

sénateurs représentant les Français établis hors de France au mois de septembre prochain. C'est la solution qui nous paraît la plus claire, la plus simple et la mieux fondée juridiquement.

Si le virus continue de circuler sur notre territoire, nous nous accordons tous sur le fait que sa progression semble maîtrisée, voire contenue et même affaiblie. Après des semaines de bilans journaliers plus terrifiants les uns que les autres, la France reprend enfin son souffle, pendant qu'une autre partie du monde continue de sombrer dans la crise sanitaire. En bouleversant l'organisation même de nos foyers, de notre manière de travailler, de consommer et de vivre, le virus a aussi perturbé le cours de notre vie démocratique. de mars dernier, près de 48 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur nouvelle équipe municipale dans les 35 000 communes qui constituent le coeur battant de notre démocratie locale. Dans 30 000 d'entre elles, le soir de la victoire d'une liste au premier tour a vu les Français rentrer ou rester chez eux pour se calfeutrer et résister à une menace rampante, invisible et meurtrière. Pour les 5 000 autres, le second tour prévu le dimanche 22 mars 2020 a été annulé le jeudi 19 mars. Nos territoires ont donc dû se préparer à affronter en première ligne une crise sanitaire sans précédent, en étant privés, pour certains, d'un exécutif local stable et établi.

Mais, à notre grande surprise, fut déposé concomitamment sur le bureau du Sénat un projet de loi organique visant à reporter les élections sénatoriales et les élections législatives partielles, sur le fondement d'un hypothétique report des élections municipales au-delà de juin 2020. Si les trois dernières années, en particulier les trois derniers mois, ont mis à rude épreuve notre calendrier parlementaire, avec des expériences gouvernementales, nous voici maintenant devant une originalité : les « projets de loi fictions

N'avons-nous pas démontré que nous étions capables de nous réunir en urgence pour prendre nos responsabilités, écrire la loi, l'amender et la voter dans l'intérêt général ? Ne l'avons-nous pas fait voilà quelques semaines à propos de l'état d'urgence sanitaire et voilà quelques mois pendant la crise des « gilets jaunes » ? N'allons-nous pas le faire une nouvelle fois la semaine prochaine, lorsque nous débattrons de la sortie de l'état d'urgence sanitaire ? Au rebours du bon sens, sénateurs et députés ont été appelés à se pencher sur des fictifs opposés, relus simultanément par chacune des chambres parlementaires, avec un énième script qui nous réunit aujourd'hui dans cet hémicycle, pour nous attacher sans prétention à compléter des dispositions de la Constitution, socle fondateur de notre République.

Au lieu de cela, nous avons passé des heures sur un texte fictif protéiforme. La commission des lois, sur l'initiative de son président, a dû siffler la mi-temps pour que, à l'issue de nos travaux, soit promulguée une loi, et non une boîte à outils législative de secours. projet de loi organique portera donc uniquement sur le cas des sénateurs représentant les Français de l'étranger, en raison de l'impossibilité matérielle d'organiser les élections consulaires dans certains pays sur lesquels déferle actuellement la vague pandémique. En commission, le Gouvernement a pu apporter des solutions sur l'ensemble des points juridiques évoqués dans la motion tendant au renvoi déposée par M. le rapporteur Philippe Bas. Ce texte

Nous sommes également satisfaits de l'adoption de l'amendement du rapporteur validant l'interprétation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique quant aux obligations déclaratives s'imposant aux parlementaires pendant la crise sanitaire.

Les sénateurs représentant les Français de l'étranger sont bien conscients de cette réalité. Le projet de loi organique que nous examinons aujourd'hui prévoyait initialement le report de l'élection

lors que l'on considère que la jurisprudence du Conseil constitutionnel l'empêche, il faut rechercher une solution permettant de se conformer aux exigences de la démocratie telles que le Conseil constitutionnel les a interprétées,

ce débat ? L'élection du président du Sénat et de l'ensemble des instances de notre assemblée est réglée par l'article 32 de la Constitution ; la désignation de nos représentants à la Cour de justice de la République est réglée par un autre article de la Constitution. Il est prévu que ces désignations ont lieu

pour un cas de force majeure et afin d'assurer le bon fonctionnement de l'expression du suffrage universel indirect, ce qui est tout de même un objectif essentiel, nous devons considérer que cela n'a pas d'incidence sur le renouvellement des instances du Sénat. D'ailleurs, les collègues dont le mandat va être prolongé, si l'on suit la demande du Gouvernement et l'avis de la commission des lois, seront des sénateurs de plein exercice au mois d'octobre prochain, représentant pleinement les Français de l'étranger et participant de manière pleine et entière à l'élection des instances du Sénat. Ce ne seront pas des demi-sénateurs pendant la prolongation de leur mandat

Évidemment, on doit apprécier le renouvellement d'un corps électoral pour chaque circonscription, c'est-à-dire le monde

Je vous remercie se pose la question suivante : que faire, à l'approche d'un renouvellement sénatorial, lorsque les grands électeurs devant élire une partie des sénateurs d'une série n'auront pas été renouvelés ?

que le Conseil d'État n'a pas pu se prononcer sur le texte dont nous débattons, puisque le Gouvernement a introduit ces dispositions par voie d'amendements

dans l'intérêt de la démocratie. En effet, il n'est pas bon que les mêmes grands électeurs désignent deux fois de suite

Je tiens quand même à préciser que la décision que nous avons à prendre ne consiste pas à supprimer jusqu'en 2021 six sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France ! Les sénateurs dont le mandat serait prolongé par la loi organique seront des sénateurs de plein exercice ; ils participeront à toutes les désignations internes au Sénat et pourront être eux-mêmes candidats à tous les postes qui seront ouverts à l'occasion du renouvellement partiel du Sénat.

qu'une assemblée prolonge le mandat de certains de ses membres est, d'une certaine façon, contradictoire avec l'idée même de la démocratie. Pour nous

En outre, cet amendement suggère que les électeurs pourraient se déplacer pour voter à l'urne dans leur pays d'accueil ou voter par procuration ou le système spécifique de remise de vote en main propre à Paris, alors que la plupart des vols ne seront peut-être pas rétablis et qu'ils ne peuvent pas voter par internet.

Qu'en sera-t-il en septembre ? Personne ne peut le savoir aujourd'hui. Comment les élus pourront-ils se déplacer dans les différents postes diplomatiques et bureaux de vote à l'étranger si cette situation perdure ? Rappelons que, pour établir une procuration, il faut de toute façon se déplacer au moins une fois. Rappelons aussi qu'il s'agit non pas d'une centaine d'électeurs, comme avant 2013, mais de près de cinq cents, répartis dans toutes les parties du monde, dont certaines sont très affectées par la crise sanitaire.

de 2014 ne vivent plus aujourd'hui dans le pays où ils étaient expatriés au moment de l'élection. Il en résulte que

de trois, de quatre ou de cinq ans. On ne peut pas faire n'importe quoi : nous sommes assujettis au respect de principes qui sont ceux de la démocratie ; nous avons juste besoin

favorables, au nom de la légitimité de notre assemblée, à ce que chacun d'entre nous soit élu par un corps électoral réellement représentatif des Français qui l'ont désigné. C'est tout de même une règle de base, il n'est même pas besoin de faire du juridisme, d'entrer dans le détail des principes constitutionnels pour l'affirmer énergiquement

revoter une loi organique pour fixer la date d'élections sénatoriales partielles, qui devraient nécessairement avoir lieu non pas dans le délai de trois mois prévu en cas de

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

confirmait l'intention que semble avoir exprimée le Président de la République à cet égard de reporter de vingt mois

projet de loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Le scrutin est ouvert.

a adopté le projet de loi organique. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

fils ou une fille puisse voter pour sa mère ou son père âgé, même quand il n'est pas inscrit sur la liste électorale de la commune. Et je ne vois pas en quoi nous courions le moindre risque de fraude. Je déploreque cela n'ait pas été rendu possible. Pour autant, j'apprécie que la majeure partie des dispositions de la proposition de loi que j'avais eu l'honneur de présenter avec mes collègues Bruno Retailleau et Hervé Marseille ait été retenue des travaux de la commission mixte paritaire. De cela, je suis très satisfait. Naturellement, nous avons écarté toutes les dispositions dont vous n'aviez plus besoin,

de cette question que nous avions à trancher, nous avons pu aussi introduire des dispositions que je trouve fort intéressantes sur les élus des Français établis hors de France. À cet égard, je tiens à saluer la proposition

mixte paritaire. Et la plupart de ces dispositions très importantes ont été accueillies avec bienveillance par nos collègues de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues élus des Français de l'étranger, vous ne rentrerez pas bredouilles à la maison Vous pourrez dire que le travail accompli, ces dernières années ou ces dernières semaines, pour faciliter la vie de ceux qui sont auprès des Français

Je me réjouis donc de ces apports et je me félicite que le Sénat ait été entendu. Cela ne signifie pas que nous ayons eu tout ce que nous souhaitions, mais nous avons obtenu beaucoup

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Président de la République l'a annoncé dimanche dernier : les élections municipales se tiendront bien, sauf exception locale, le 28 juin prochain. Nous regrettons que les conditions sanitaires en Guyane ne permettent pas la tenue d'un second tour. Tout doit être fait pour que la situation s'y améliore rapidement. Même s'il faut rester prudent, l'épidémie semble toujours sous contrôle en métropole, comme l'indiquait le comité scientifique au début du mois. Nous nous réjouissons que la situation sanitaire se soit améliorée. Sans oublier les morts et les efforts remarquables des professionnels de santé, dans son adresse aux Français, le chef de l'État a insisté sur le fait que notre pays a tenu bon. a tenu bon. Une fois encore, nous saluons l'engagement du personnel médical. De plus, nous nous réjouissons que le Parlement se soit montré à la hauteur et que les deux chambres aient su travailler en si bonne intelligence. La gestion de la crise doit aussi beaucoup à l'engagement et au travail des élus de terrain, qui sont la colonne vertébrale de notre République. Ils ont beaucoup fait, et pas seulement durant cette crise. Néanmoins, ils doivent pouvoir agir avec une pleine légitimité. Au total, quelque 16,5 millions de Français attendent encore le second tour qui permettra la formation de leur conseil municipal.

Ceux qui se déplaceront pourront, quant à eux, se faire remettre un masque lors de leur arrivée au bureau de vote. Toutes ces mesures concourent à ce que les électeurs puissent voter sans risque pour leur santé. Nous espérons ainsi que la participation au second tour sera bien plus forte que le 15 mars dernier. Si les conditions sanitaires s'améliorent globalement en France, il n'en va pas de même dans le reste du monde : les chiffres des contaminations continuent d'augmenter à l'échelle mondiale. Comme on ne peut pas garantir que les scrutins se dérouleront dans des conditions satisfaisantes, il nous semble plus sage de reporter les élections consulaires au mois de mai 2021. Au surplus, tant que la situation n'est pas totalement revenue à la normale, nous paraît préférable que les assemblées locales puissent continuer à fonctionner selon des procédures plus simples et plus souples. Doucement, la France reprend vie. Nous allons devoir vivre encore au moins plusieurs mois avec le virus. Il nous faut rester unis, comme nous l'étions au plus fort de la crise sanitaire, pour permettre à notre pays de retrouver une activité normale. Ce texte de compromis y concourt : c'est pourquoi le groupe Les Indépendants le votera. La parole est à M.

l'ont rappelé -, le texte adopté en commission mixte paritaire traite principalement de deux sujets : premièrement, le report des élections consulaires ; deuxièmement, les aménagements permettant de faciliter le vote de nos concitoyens les plus fragiles. J'évoquerai brièvement ces deux aspects. Tout d'abord, concernant les élections consulaires, on comprend aisément que la problématique était bien différente de l'organisation d'un second tour sur le territoire national. L'épidémie connaît diverses évolutions à travers le monde, certaines régions pouvant connaître des pics ou des rebonds. Les déplacements vers les bureaux de vote se seraient révélés d'autant plus difficiles que les électeurs doivent parfois parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour accomplir leur devoir électoral.

Les travaux de nos deux assemblées ont également permis de créer un dispositif particulier en cas de cluster identifié d'ici au 28 juin prochain. En cas de besoin, l'article 5 du projet de loi permettrait à l'exécutif d'annuler le scrutin dans un nombre limité de communes qui C'est la situation sanitaire en Guyane et à Mayotte que nous avions en tête lors de nos débats. L'actualité récente nous montre que ces craintes étaient malheureusement justifiées dans le cas du département de la Guyane. concernant le régime des procurations, nous nous félicitons que la voix du Sénat ait été entendue. Chaque mandataire pourra bien disposer de deux procurations, et les mandants pourront

Enfin, le groupe Union Centriste salue le fait que la commission mixte paritaire ait validé plusieurs mesures défendues par certains de ses membres et visant à faciliter le fonctionnement des assemblées locales. Par exemple, il était nécessaire d'adapter le calendrier de renouvellement de certaines instances, comme les comités des syndicats mixtes. En vertu du texte

Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en dépit des conditions particulières dans lesquelles nous sommes tenus de légiférer, et qui sont d'ailleurs l'objet même de la plupart des textes en discussion, le dialogue parlementaire a, une nouvelle fois, montré toutes ses vertus : c'est encore encore plus vrai à l'heure du recours massif aux ordonnances et de la généralisation de la procédure accélérée. La qualité de la loi en dépend. L'accord trouvé en commission mixte paritaire en atteste. Le groupe du RDSE se réjouit de retrouver dans ce projet de loi l'essentiel de la proposition de loi à laquelle travaillait le Sénat pour faciliter le recours à la procuration. Sur ce sujet, les élus de mon groupe avaient fait de nombreuses propositions. Cette exigence, aussi bien démocratique que sanitaire, devait être satisfaite. Il appartient désormais au Gouvernement de placer l'administration dans les meilleures conditions, pour rendre effectives les mesures que nous nous apprêtons à voter. Nous savons les qualités et le dévouement de nos fonctionnaires et nous ne doutons pas qu'ils sauront se mobiliser, afin de recueillir les procurations des électeurs dans ces circonstances si particulières.

Le régime dérogatoire prévu pour ces communes l'illustre, avec un délai de quatre semaines laissé pour organiser de nouvelles élections après une éventuelle annulation. À cet égard, nous avons une pensée particulière pour nos compatriotes guyanais et mahorais. Les nombreuses clarifications, notamment temporelles, dans les aménagements transitoires du droit des collectivités territoriales, rendues nécessaires par l'épidémie de Covid-19, sont, elles aussi, les bienvenues. Il en va ainsi des modalités de réunion des organes délibérants, de partage des compétences en leur sein et d'organisation des exécutifs locaux. Les précisions relatives aux élections des désormais « conseillers des Français de l'étranger » s'accompagnent d'un statut propre à leur offrir de meilleures conditions d'exercice de leurs fonctions. Elles sont donc autant de moyens de susciter des vocations. élus bénéficieront d'aménagements dans leurs rapports avec leur employeur et de la garantie que leurs absences professionnelles dues à leurs obligations de conseillers ne diminueront pas la durée de leurs congés payés ou leurs droits aux prestations sociales.

notamment du fait de la désignation tardive des délégués municipaux et de leurs suppléants, qui n'ira pas sans créer de la complexité pour nombre de candidats. Au-delà de cet aspect particulier, il reste une question qui transcende toutes ces élections, et dont nous allons entendre parler durant plusieurs années. Il s'agit des conditions dans lesquelles se sont déroulés, et se dérouleront demain, les scrutins dont la pleine expression se trouve manifestement affectée. Les élus désignés par les urnes en mars et en juin 2020 auront pourtant de lourdes responsabilités à assumer,

Aux questions qui se poseront demain, nul ne peut encore apporter de réponse certaine ; mais les conclusions dont nous discutons aujourd'hui, sur lesquelles se sont accordées les deux assemblées, sont le fruit d'une méthode que nous pouvons défendre. Dans cette situation éprouvante, souhaitons que les leçons que nous pouvons légitimement tirer du travail parlementaire soient prolongées. Si le dialogue institutionnel,

Mon propos n'a pas changé et, au risque d'être quelque peu redondant aujourd'hui, je tiens à déclarer que nous soutenons le texte issu de la commission mixte paritaire, car il est à la hauteur des enjeux démocratiques que revêt le scrutin du 28 juin Je tiens à souligner la très grande réactivité du Sénat, laquelle est constante depuis le début de la crise sanitaire. Nous pouvons collectivement être fiers d'avoir fait preuve d'efficacité dans l'examen de ce texte, d'autant que nous n'avons pas sacrifié notre exigence technique et politique sur l'autel de la productivité légistique.

Ils ne m'empêcheront pas de penser que l'efficacité de notre travail et sa rigoureuse qualité sont les deux marques de fabrique de notre institution. Les solutions proposées par ce texte font, elles aussi, preuve d'adaptabilité et répondent aux enjeux d'une situation inédite complexe.

Un second exemple illustre l'adaptabilité de notre travail parlementaire : la différenciation proposée par ce projet de loi comme réponse à la crise. C'est bien une forme de différenciation inédite que permet l'article 5 de ce projet de loi : une différenciation électorale. En effet, le Gouvernement a proposé au Parlement de permettre le report du scrutin dans les communes constituant un cluster. Quelle meilleure réponse pouvions-nous apporter pour exprimer notre volonté de faire face aux réalités sanitaires locales ?

Il permet également à ceux qui, en raison de l'épidémie, ne pourront pas se déplacer, de solliciter la venue des autorités à leur domicile, pour établir et recueillir leur procuration sans avoir à fournir de justificatif, par exemple médical. Cette solution est en tout point équilibrée. Elle permettra au plus grand nombre de voter le 28 juin et elle est techniquement envisageable dans un délai court, sans risque de fraude. Ensuite, je pense à nos candidats, à nos futurs élus, d'entre eux qui s'impatientent et qui méritent la plus grande clarté. La clarification de la date de leur entrée en fonction pour les communes où le scrutin serait reporté, l'allongement des délais de recours, ou encore la dématérialisation du dépôt de candidatures pour les élections consulaires sont autant de mesures attendues et de clarifications nécessaires à la bonne reprise de notre vie démocratique. je pense aux collectivités territoriales. Les allègements permis par ce texte, visant à faciliter leur vie institutionnelle en période d'épidémie et de reprise, répondent à une demande forte de leur part. Extension de l'allègement des règles de quorum et de pouvoir dans les assemblées délibérantes ; fixation rétroactive des indemnités, au plus tard le 30 septembre prochain ; possibilité donnée au conseil municipal de se réunir en tout lieu ; limitation possible du public aux réunions du conseil municipal

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le feuilleton des élections municipales, même si le présent texte est censé en arranger au mieux les contours, ne semble malheureusement pas terminé. le ministère de l'intérieur a annoncé l'annulation du second tour et le report des élections municipales en Guyane, faisant déjà application du fameux article 5 de ce projet de loi, pourtant

Nous approuvons les mesures visant à favoriser la participation par la possibilité d'établir deux procurations et celles destinées à sécuriser les opérations et les bureaux de vote avec le soutien financier total de l'État. Elles vont dans le bon sens, même si leur adoption tardive- le scrutin aura lieu dans dix jours ... -révèle encore une fois la confusion dans laquelle le Gouvernement a géré l'organisation des élections municipales. Les apports du Sénat permettant aux instances locales de continuer à fonctionner de manière sereine et adaptée à la situation sanitaire, toujours instable, et aux conséquences du report du second tour sont également bienvenus.

En déroulant toutes ces mesures, nous touchons du doigt les conséquences multiples de cette gestion, disons chaotique, des élections municipales et de leur maintien en mars dernier. Un constat qui nous amène à questionner la constitutionnalité et la solidité juridique des solutions proposées le casse-tête n'est pas fini, puisque, lorsque nous aurons traité des sénateurs représentants les Français de l'étranger, il nous faudra trouver une solution aussi pour les sénateurs renouvelables de Guyane, alors que sept communes guyanaises devront tenir deux tours de scrutin d'ici au Nous sommes dans une situation inédite, dont la difficulté tient aux incertitudes de l'épidémie qui affecte notre vie quotidienne depuis plusieurs mois, mais aussi à l'instabilité sociale et économique qui en découle. Ce contexte pèse très fortement sur le second tour. un sondage de l'Ifop paru cette semaine, seulement 38 % des Français concernés iraient voter le 28 juin prochain. De fait, l'état d'esprit de nos concitoyennes et concitoyens n'est pas d'aller aux urnes, et cette campagne électorale inédite, sans contact, malmène la démocratie encore confinée. Cet étrange climat se nourrit également de l'actualité internationale. Ajoutons-y les craintes renforcées par la récente étude de chercheurs de Clermont-Ferrand liant premier tour des élections municipales et taux de mortalité du Covid-19, et nous avons là tous les ingrédients d'une abstention massive, préjudiciable à la démocratie. Bien que ce texte soit un moindre mal, nous nous abstiendrons, en cohérence avec notre position sur la gestion de ces élections par l'exécutif, une gestion qui a provoqué l'instabilité Le droit pour les citoyens d'élire leurs représentants, le respect du suffrage universel et la tenue d'élections sont au fondement de notre démocratie : ils ne sauraient souffrir d'hésitations, d'atermoiements ou de petits calculs. Je songe évidemment à ce que nous apprenons de la négociation que tenterait Emmanuel Macron pour reporter les élections régionales après les présidentielles, en échange de soutiens financiers aux régions.

Deromedi. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, au terme de l'ordre du jour de cette semaine, nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation du second tour des élections municipales et au report des élections consulaires. Ce texte, déposé à la fin du mois dernier devant l'Assemblée nationale, visait initialement à permettre l'annulation éventuelle du second tour des municipales, tout en assurant le report, qui est quant à lui certain, des élections consulaires. il a fortement évolué dans la bonne direction, à la faveur du travail réalisé par nos deux assemblées, en particulier par le rapporteur du Sénat, le président Philippe Bas. Nous avions abordé ce projet de loi avec une certaine circonspection. De fait, comme le rapporteur en a habilement fait la démonstration en séance la semaine dernière, voter une loi en grande partie virtuelle posait de multiples problèmes, le moindre n'étant pas celui de la constitutionnalité de telles dispositions. À d'autres égards, notre commission avait considéré que le texte demeurait trop muet sur les questions tenant aux aménagements de l'organisation concrète de l'élection. de cette élection est de plus en plus improbable ; nous avons pu lire, en début de semaine, l'avis du conseil scientifique confirmant son évaluation précédente sur ce sujet. il aurait été incompréhensible de s'en tenir à l'unique mesure prévue par les députés, les doubles procurations, reprenant au demeurant une disposition proposée et votée par le Sénat bien auparavant. C'est donc avec satisfaction que je constate, au nom de mon groupe, que les équilibres essentiels votés par notre assemblée sont respectés dans le texte adopté par la commission mixte paritaire, à laquelle j'ai participé. Il a été possible de convaincre les députés du bien-fondé de nos positions et de faire de ce projet de loi un outil au service du bon déroulement d'un processus électoral essentiel sur le plan démocratique, mais malheureusement interrompu par l'épidémie.

reviens pas. Je salue aussi le maintien dans le projet de loi des dispositions relatives aux procurations électorales et au bon déroulement des élections de juin 2020, qui trouvent leurs origines dans la proposition de loi des présidents Bas, Retailleau et Marseille du 22 mai dernier.

Pour ce scrutin uniquement, ces dispositions permettront à chaque mandataire de disposer de deux procurations, doublant ainsi les possibilités actuellement prévues par la loi. En outre, les personnes les plus exposées pourront faire établir des procurations depuis chez elles, dans un cadre juridique simplifié. Enfin, l'article 1 garantira le financement par l'État de la mise à disposition dans les bureaux de vote d'équipements de protection, à destination aussi bien de leurs membres que des électeurs. Outre les mesures relatives au déroulement du prochain scrutin,

L'article 5, qui maintient la possibilité d'annuler la tenue du scrutin dans certaines communes, a aussi été conservé. Compte tenu de la situation très spécifique dans les territoires où le virus circule encore fortement et où des clusterspersistent, notamment en Guyane et à Mayotte, cette mesure nous a semblé suffisamment proportionnée et encadrée pour être maintenue. Enfin, permettez-moi de revenir sur certaines dispositions du texte final qui ont tout particulièrement retenu mon attention, ainsi que celle de mes collègues représentant les Français établis hors de France.

était nécessaire, car nous avons pu constater dans de nombreux pays que l'évolution de l'épidémie demeure préoccupante. La mobilité des personnes y est encore limitée, et les vies de nos compatriotes ont été désorganisées. Il était impératif de laisser à la situation le temps nécessaire pour se clarifier et permettre un bon déroulement du processus démocratique, dans des conditions sanitaires satisfaisantes. sanitaires satisfaisantes. Le Sénat ne s'est pas borné à affiner la question du report de cette élection, ni même à ajuster les conditions de déroulement de celle-ci. Il a aussi adopté un nombre important de dispositions supplémentaires relatives aux Français de l'étranger. mesures reprennent certaines des avancées que notre assemblée avait déjà votées à l'occasion de plusieurs propositions de loi dont j'avais eu l'honneur d'être le rapporteur, en janvier 2019, puis en mai dernier. mai dernier. Ces avancées portent notamment sur les garanties en termes d'autorisation d'absence pour assister aux réunions, de prise en charge des frais de déplacement et de reconnaissance protocolaire des élus des Français de l'étranger. Sur un plan pratique, la loi comportera aussi des dispositions de simplification de la procédure de dépôt des déclarations de candidature aux élections consulaires. Par ailleurs, nous espérons que l'introduction dans la loi d'une demande de rapport du Gouvernement à l'Assemblée des Français de l'étranger et la consultation obligatoire de cette assemblée sur la mise en place du vote électronique permettront de pérenniser ce mode de scrutin. Enfin, je salue l'entrée en vigueur prochaine de la nouvelle dénomination souhaitée par les conseillers consulaires : devenus conseillers des Français de l'étranger, ils seront mieux identifiés par nos compatriotes. En particulier grâce aux travaux du Sénat, ce projet de loi permettra d'apporter des garanties et assurances fortes, en vue de l'organisation tant des élections municipales que des élections consulaires.

lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.